Les infrastructures de notre pays- les réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux -doivent faire l'objet d'une vision claire, et les projets engagés Chaque projet engagé, par exemple l'aménagement d'un tronçon sur un axe du réseau routier national, s'inscrit dans une vision d'aménagement de plus long terme. Cet amendement vise à contribuer à rendre effective l'exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics, qui découle de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

mais aussi de faciliter et de décarboner le transport au quotidien des habitants. Par ailleurs, développer la mobilité au moyen d'une liaison tram-train, lorsque cela est possible, permet le désenclavement des territoires des transports décarbonés répond au double enjeu de l'attractivité des territoires et de la réduction de la pollution. Favoriser les transports décarbonés à un coût abordable pour l'usager, grâce aux transports guidés, tel est l'objet de cet amendement.

afin de respecter l'équilibre nécessaire entre, d'une part, les besoins en déplacement des personnes et des marchandises et, d'autre part, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le secteur des transports. Ses dispositions s'intègrent donc parfaitement dans les priorités que vous avez données,

dit, ces propositions posent des difficultés. Je ne les citerai pas toutes, mais la proposition qui vise à subordonner tout projet de construction, d'extension ou de modification d'infrastructure à l'impossibilité de pourvoir aux

un article qui engage les pouvoirs publics à maintenir et à développer les équipements et réseaux existants, notamment dans le domaine ferroviaire, afin d'éviter, par exemple, la dégradation des trains d'équilibre du territoire ou des trains d'aménagement du territoire, ou encore la fermeture de gares de TGV. À titre d'exemple, cela a été évoqué précédemment, sur la ligne Lyria, on envisage une modification du cadencement des TGV, ce qui pourrait infléchir la fréquentation de certaines gares, dont la desserte serait

: depuis 2011, les transporteurs sont contraints d'informer leur donneur d'ordre de la quantité de gaz à effet de serre produite par le transport.

a décidé de transporter ses voitures sur des camions parce que le transport routier était devenu plus compétitif de quelques euros que le transport par barges, sur la Seine. Si un tel donneur d'ordre

De plus, cela a été souligné dans de nombreux rapports, cette formule conduit à un renoncement, par la puissance publique, à sa compétence de maîtrise d'ouvrage. Cela entraîne une

matière. Sur le papier, ces montages sont censés optimiser le partage des risques entre le public et le privé et mobiliser de nouvelles ressources financières privées, afin de réaliser de grands projets d'utilité nationale.

Même avis.

de la commission ? Nous sommes tous sensibles à cette question. Le Gouvernement a déjà rendu un rapport identifiant les ponts nécessitant des interventions pour renforcer leur sécurité.

Quoi qu'il en soit, nous avons anticipé et veillé, dans le rapport annexé, à ce que les investissements de l'État dans les infrastructures permettent de renforcer cette sécurité. Nous avons prévu des budgets spécifiques sur cette question dans le texte.

que, comme nous le savons, ces rapports ne sont pas toujours fournis. Ce que je dis est purement factuel, madame la ministre. Chaque année, le bilan d'application des lois fait apparaître, pas seulement dans votre ministère, mais de manière générale, un taux de remise des rapports demandés par le Parlement extrêmement peu satisfaisant. je ne peux qu'aller dans le sens de la demande de retrait formulée par M. le rapporteur et Mme la ministre.

que le droit à la mobilité est antinomique, et même contradictoire, avec le maintien de ce pacte ferroviaire. Comme nous l'avions défendu à l'époque, nous considérons que cette loi est mortifère pour le service public ferroviaire et donc pour le droit à la mobilité affirmé par l'article 1 de ce projet de loi d'orientation des mobilités. En effet, en prévoyant l'ouverture à la concurrence, le changement de statut de l'entreprise publique, la filialisation des activités et la fin du statut des cheminots, cette loi porte les germes d'une privatisation future de l'entreprise nationale, qui sera préjudiciable aux usagers et au service public. Elle ouvre également le risque d'une balkanisation de l'offre, de l'abandon d'un certain nombre de lignes, comme le comme le confirment des annonces récentes, et d'une désorganisation de l'entreprise historique, en mettant fin à la péréquation nationale entre les différentes activités de l'opérateur public. S'appuyant sur le rapport Spinetta qui n'a toujours pas été renié par le Gouvernement, ce texte prépare la désertification des territoires par la réduction

où l'on socialise les pertes et où l'on privatise les profits. C'est même le fil rouge de l'action de votre gouvernement : donner au privé les secteurs rentables- autoroutes, Aéroports de Paris -, de Paris -, pour ne parler que du secteur des transports. Pour le reste, vous proposez, selon vos propres mots, des solutions de mobilité, mais le service public et l'offre structurelle de masse ne sont plus assurés. À notre sens, une telle conception du système national de transport ferroviaire met à mal le droit à la mobilité et le maillage du territoire par les réseaux ferroviaires en soumettant la présence d'une offre de transport à une rentabilité suffisante pour les opérateurs privés. Pour ces raisons, nous proposons d'abroger

du Gouvernement ? En effet, on ne va pas refaire le débat sur la loi ferroviaire. Je ne suis d'accord avec à peu près aucun des points que vous avez évoqués. Je rappelle que l'objectif de cette loi, c'est bien un meilleur service au meilleur coût, avec une ouverture à la concurrence,

Je rappelle que ce nouveau pacte ferroviaire s'accompagne d'un effort considérable de la Nation en faveur du ferroviaire, avec une augmentation de 50

tout. Beaucoup de nos concitoyens, aujourd'hui, n'ont pas d'autre solution que la voiture. La loi dont nous débattons aujourd'hui doit donc permettre de compléter les offres ferroviaires par d'autres offres

Cela nécessite évidemment de revenir sur les modalités de l'ouverture à la concurrence, qui a laissé la main invisible du marché organiser, ou plutôt désorganiser, ce secteur d'activité. Résultat

de plus en plus. En tant qu'élue de la Seine-Maritime, je ne peux m'empêcher d'évoquer le port du Havre, le plus important en France pour le trafic de containers. Sachez que moins de 5 % des marchandises qui transitent par le port du Havre sont aujourd'hui acheminées par le rail.

sur le nouveau pacte ferroviaire, nous avons remis à plat les trajectoires de péages, qui prévoyaient une augmentation de 8 % à 10 % par an des péages de fret pour les stabiliser au niveau de l'inflation. Nous soutenons le report modal avec une aide au transport combiné de 27 millions d'euros sur cinq ans et remettons en état les lignes capillaires pour permettre la logistique du dernier kilomètre dans les territoires. Nous avons également demandé à SNCF-Réseau de consacrer 20 millions d'euros par an pendant trois ans pour la remise en état des voies de service. La programmation, dont nous venons de débattre, prévoit aussi des moyens importants pour améliorer les grands itinéraires, en particulier ceux qui desservent nos ports. S'agissant du port du Havre,

la continuité de service est un enjeu majeur pour les chargeurs. Or les mouvements que l'on a connus l'an dernier ne vont pas dans le sens d'une relance du fret ferroviaire. L'avis est défavorable. La parole est

Gontard, sur l'article. L'article 1 de ce texte a deux objets. Il transforme le droit au transport en droit à la mobilité, et il organise la gouvernance de cette compétence pour l'inscrire dans le couple formé par l'intercommunalité et la région, qui deviennent les autorités organisatrices de la mobilité. Nous nous sommes déjà exprimés sur le changement de terminologie, qui, sous couvert d'embrasser mieux une réalité diverse et évolutive des mobilités, rompt en fait avec une certaine vision du système de transport, fondé sur un service public et des opérateurs publics. Il est question ici non pas d'offre de transport, mais de solutions de mobilité, qui deviendront,, l'argument pour ne pas investir dans du transport collectif. Cette vision n'est, hélas, ni moderne ni écologiste, puisqu'elle fait de la route le principal support des offres de transport. Elle ne répond pas aux enjeux, car elle passe totalement à côté du besoin de transport de masse que représentent les transports en commun. Si nous partageons l'idée qu'il faut s'appuyer et favoriser l'ensemble des solutions alternatives à la voiture individuelle, en zone rurale, où l'offre de transport public est faible, cet objectif ne peut pas nous faire perdre de vue que toutes les mobilités ne se valent pas, qu'elles ne remplissent pas toutes la même fonction. Faire du covoiturage l'alpha et l'oméga de toute politique des transports n'est pas une bonne idée, car, en creux, comme avec les cars Macron, cela discrédite toute idée de la nécessité d'un service public, porté par des opérateurs publics, tourné non pas vers les axes où il y a de la demande, mais sur l'existence d'un droit. Nous sommes donc circonspects et inquiets face à ces évolutions. En ce qui concerne la gouvernance, reconnaissons d'abord une volonté, celle de couvrir l'ensemble des territoires d'autorités organisatrices. Pour cela, toutes les intercommunalités deviennent autorités organisatrices, avec un mécanisme de transfert de compétence obligatoire des communes. Vous le savez, nous n'aimons pas beaucoup ces injonctions aux communes, mais c'est un autre débat. Nous espérons simplement, avec l'achèvement de la carte intercommunale, qui ne correspond pas toujours à des intercommunalités choisies, que ces mécanismes ne vont pas contribuer à créer de nouvelles zones blanches. Sur le fond, nous partageons cette volonté de lutter contre l'assignation à résidence, encore faut-il que les nouvelles autorités organisatrices aient concrètement les moyens de développer des offres de transport, mais nous y reviendrons avec la question du versement mobilité, au prochain article. La Piednoir, sur l'article. Le projet LOM se fixe comme objectif d'améliorer la gouvernance des mobilités avec la couverture de tout le territoire par une autorité organisatrice de la mobilité, AOM, et une coordination des compétences entre ces autorités. Il donne la primauté aux intercommunalités pour exercer, ou non, la compétence mobilité. À défaut, les régions devront se substituer à elles, ce qui conduira, selon moi, à un morcellement de l'exercice des compétences entre territoires ayant choisi de s'en emparer et ceux qui auront préféré laisser la région s'en charger. Plusieurs points appellent notre vigilance. D'abord, il y a un risque de confusions pour les usagers et les élus locaux. Issu de la loi NOTRe, le transfert des lignes interurbaines et scolaires des départements aux régions n'est encore ni digéré ni stabilisé. Les conséquences en matière de continuité de service, de tarification ou de gestion avec les autorités organisatrices de second rang ne favorisent pas toujours une bonne lisibilité ni une proximité satisfaisante pour les usagers de ces services et pour les élus, qui ont besoin de temps et de stabilité. nous pointons un risque de perte d'efficience des services de transport. Le périmètre pertinent des services de transport ne se limite pas toujours aux frontières des intercommunalités qui prendront la compétence mobilité. Nous devrons veiller à ce que la continuité des services soit garantie au-delà des limites territoriales des nouvelles AOM, non seulement pour le transport lui-même, mais aussi pour la tarification, la billettique ou l'information des usagers. Assurons-nous que les régions disposeront bien des prérogatives leur permettant d'exercer effectivement le rôle de chef de file que ce projet de loi leur confie. Il n'est pas assuré que ce soit le cas en l'état.

qui attendent que de nouveaux services performants de mobilité se mettent en place. Cela requiert un financement, dont les intercommunalités sous-estiment d'ailleurs souvent le niveau, et que la perception d'un versement mobilité au taux maximal de 0,3 % ne permettra pas de couvrir, dans les zones rurales, où le tissu d'entreprises de plus de onze salariés est souvent fragile. l'article. Vous nous proposez un article extrêmement important, qui vise, ni plus ni moins, à redéfinir le code des transports en substituant la notion de mobilités à celle de transports. J'insisterai sur la notion de droit à la mobilité durable pour tous.

aérien se sont closes la semaine dernière, et nous n'avons pas de possibilité d'intervenir sur ce sujet. Le transport des marchandises, qui vient d'être évoqué, est aussi un parent pauvre de ce texte. Je le regrette

habitants de ces derniers étant plus ou moins condamnés à l'utilisation de la voiture individuelle si nous n'arrivons pas à inverser la tendance. Je conclus sur la notion d'enclavement. Les territoires enclavés sont vastes. Il y a non seulement les territoires ruraux, d'où je viens, mais également le périurbain. Il arrive qu'il y ait des poches enclavées à l'intérieur des villes

important. La crise que connaît notre pays depuis quatre mois montre à quel point les différences d'accès à la mobilité sont aujourd'hui source d'inégalités entre nos concitoyens et nos territoires. En effet, les grandes agglomérations ont bien souvent mis en place des transports collectifs performants, qui constituent une réponse adaptée en milieu urbain. En revanche, peu de communes ou de communautés de communes ont pris en main la compétence d'organisation de la mobilité. Face à ce constat, l'article 1 vise à faciliter

des formes différentes selon les territoires. Aussi, l'article clarifie les différentes missions des autorités organisatrices

de trouver le bon acteur à même d'exercer la compétence dans un territoire, selon un principe de subsidiarité, qui permet à la région d'intervenir si l'intercommunalité ne se sent pas en situation de le faire, et de coordination

Je n'avais pas prévu d'intervenir à ce stade, mais, puisque Mme la ministre a souhaité faire une déclaration liminaire sur cet article, je veux répondre rapidement.

Nous partageons votre ambition de passer du droit au transport au droit aux mobilités, et à toutes les mobilités, pour tous. Pourquoi cette proposition d'intégrer l'adverbe « verticalement » à cette définition de la mobilité ?

Pas d'ascenseur, c'est moins, voire plus du tout de mobilité et d'autonomie ! C'est moins de lien social ! C'est l'isolement ! Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce sujet ! Nous avons évoqué hier le transport

La sédentarité, vous le savez, est l'un des principaux maux de notre époque. Elle favorise le développement de facteurs de risques cardiovasculaires, diabète, cholestérol trop élevé, obésité ... ... Elle favorise tous les troubles musculo-squelettiques, mal de dos, de cou, d'épaule, qui sont responsables d'un grand nombre d'arrêts de travail ou sont, du moins, responsables du mal-être.

Les mobilités actives, qui constituent en effet un enjeu majeur de santé publique, doivent, à ce titre, faire l'objet d'un droit spécifique. Il ne peut exister aucun obstacle structurel à la volonté de nos concitoyens de se déplacer à pied ou à vélo. Plus de 60 % des trajets de moins de un kilomètre sont effectués en voiture, particulièrement en zone urbaine. Il est indispensable de faire évoluer les mentalités, mais également de s'assurer que toutes les infrastructures routières permettent une pratique sécurisée et agréable du vélo. L'urgence climatique et les objectifs fixés par l'accord de Paris nous obligent à repenser en profondeur notre rapport à la mobilité et aux modes de déplacement. Toute personne devrait se voir reconnaître un droit à la mobilité active lui permettant d'effectuer tous ses déplacements sur de courtes distances, dans des conditions sécurisées, bien sûr. Tel est l'objet de cet amendement, qui inscrit la lutte contre la sédentarité dans les dispositions générales du code des transports. C'est le parti

Par ailleurs, la programmation des infrastructures comprend un objectif de désenclavement. Que l'on garantisse à chacun la faculté de se déplacer, en tenant compte, le cas échéant, de son handicap, est un objectif essentiel, que nous partageons tous. Ajouter la « lutte contre la sédentarité » ne me semble pas opportun, car le sens n'est pas très clair lutte-t-on contre celles et ceux qui ne souhaiteraient pas se déplacer ? Cela donne une dimension « prescriptive » à la mobilité, avec une forme d'injonction à bouger. J'ai, comme certains, l'habitude de dire qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux ! La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. Quel est l'avis du Gouvernement du Gouvernement ? Je considère ces deux amendements identiques comme des amendements d'appel, qui sont déjà satisfaits non seulement par le droit, mais aussi par les engagements du Gouvernement.

que l'État soutient la réalisation d'infrastructures cyclables -favoriser la réalisation d'infrastructures cyclables, y compris en supprimant, le cas échéant, les discontinuités importantes qui peuvent exister. Je considère que le projet de loi qui vous est présenté comporte de nombreuses dispositions en faveur des mobilités actives. Votre amendement me semble satisfait et je vous propose de le retirer. À défaut, l'avis sera défavorable.

être soulignée. Je souscris donc tout à fait à l'amendement déposé, qui me paraît important pour les zones de montagne et les zones insulaires.

du Gouvernement ? Je pense qu'on peut en effet énumérer les diversités des situations dans nos territoires. On pourrait évoquer le monde rural, on pourrait aussi évoquer les zones périurbaines

celui de laisser de côté des territoires qui méritent aussi une attention particulière en termes de désenclavement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de votre assemblée.

présenter l'amendement n° 641 rectifié. Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs de la programmation des infrastructures l'importance du désenclavement pour les massifs de montagne qui en sont particulièrement affectés et l'amélioration de la mobilité quotidienne à l'intérieur des massifs

Lurel. Il s'agit de prendre en compte les enjeux de la continuité territoriale dans la programmation des

? Cet ajout de la continuité territoriale nous semble pertinent pour mieux répondre aux problématiques des territoires ultramarins en matière de déplacement. Avis favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? L'article 1111-3 du code des transports précise déjà que la programmation des infrastructures prend en compte les enjeux de désenclavement et d'aménagement du territoire. Il va de soi que la continuité territoriale, qui vise à compenser les difficultés

Mme Christine Lanfranchi Dorgal. Cet amendement a pour objet d'ajouter aux objectifs de la programmation des infrastructures la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique, la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Le secteur des transports constitue un secteur stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, d'une part, mais aussi pour limiter l'appauvrissement de la biodiversité, d'autre part. Le changement climatique et la pollution ont un impact direct sur cet appauvrissement du monde animal et végétal, qualifié de « sixième extinction » par les scientifiques. En vue de répondre durablement aux problématiques de gestion des espaces naturels, préservation et restauration de la biodiversité dans les territoires, il est indispensable d'agir sur les mobilités et d'intégrer ces enjeux à la programmation des infrastructures.

nous estimons que le développement de solutions complémentaires à une offre actuellement défaillante et insuffisante, telles que l'autopartage ou le covoiturage, doit rester une offre complémentaire et non une offre de substitution. En effet, elle doit non pas constituer une alternative à des services de transport public, mais, bien au contraire, se placer en stricte complémentarité pour compléter l'offre publique organisée sous la forme d'un service public. Or la rédaction de cet article, contrairement à la rédaction actuelle du code des transports, permet de remplacer l'existence d'un service public de transport par une « solution de mobilité Cette évolution nous semble porter le risque de voir diminuer une offre de service public déjà extrêmement limitée. Nous préférons donc une formule plus inclusive qui permet de placer le service public et les solutions de mobilité en complémentarité plutôt qu'en concurrence.

en prenant en considération les seuls services de transport public réguliers, on a laissé beaucoup de nos concitoyens sans solutions de mobilité.

une nouvelle rédaction de l'article L. 1111-3 du code des transports concernant certains objectifs de la programmation des infrastructures.

Nous estimons que la question des mobilités doit être traitée avec pour objectif la réduction de la fracture territoriale, en apportant des solutions concrètes, adaptées aux besoins locaux et issues d'une concertation élargie avec ensemble des collectivités locales. Il nous semble dès lors nécessaire que la programmation des infrastructures et le déploiement de l'offre de mobilité puissent faire l'objet d'un débat avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées. Tel est le sens de cet amendement.

concernés par la mobilité dans chaque territoire. C'est notamment la vocation des bassins de mobilité, des contrats opérationnels de mobilité, du comité des partenaires et des évolutions proposées

Cet amendement fixe un nouvel objectif de désenclavement à l'horizon de 2025, sur le modèle de l'article 17 de la loi du 4 février 1995 d'orientation

logistique. Cet amendement a pour objet de créer un observatoire national de la mobilité des marchandises ; c'est d'ailleurs prévu par la stratégie France Logistique 2025. Cet organisme, en préfiguration depuis trois ans, tarde à voir le jour. Or une évaluation de l'activité logistique par une entité indépendante serait utile aux collectivités locales dans l'élaboration et le suivi de leurs stratégies en matière de marchandises et aux professionnels du secteur dans l'exercice de leur activité. Il est proposé d'inscrire dans la loi cet observatoire, dont les modalités précises d'organisation seront définies par un décret en Conseil d'État. Les rémunérations et frais de fonctionnement sont à préciser,

France Logistique 2025 prévoit de mettre en place les outils d'observation des activités et services logistiques. Mais la mission de préfiguration pilotée par M. Savy a exclu la création d'une entité indépendante au profit d'une mise en réseau des sources de données. Comme l'a évoqué M. le rapporteur, la mission confiée par le Gouvernement à MM. Daher et Hémar sur l'amélioration de la compétitivité de la logistique en France doit permettre d'identifier les outils d'observation adéquats, en particulier sur la mesure de la performance. La conception et la mise en réseau des outils d'observation seront donc finalisées à la suite de la mission, en étroite relation avec les acteurs professionnels, notamment ceux qui disposent des données concernées. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

collectivités soient à cheval sur le même comité de massif. Il est absolument nécessaire d'avoir une cohérence territoriale pour la politique de mobilité à l'intérieur de ces massifs. Tel est l'esprit de cet amendement.

l'avis de la commission ? Ces trois amendements identiques visent à réaffirmer le principe de prise en compte de la diversité des besoins des territoires et de développement de solutions adaptées équitables dans l'exercice des missions de service public en matière de transports

Or la rédaction actuelle de l'article 1 laisse subsister quelques dispositions qui risquent d'aboutir à une situation contraire à l'objectif initial, c'est-à-dire au maintien de territoires où la lisibilité des offres de mobilité serait mise à mal. mal. Cet amendement a donc pour objet de remédier à de telles incohérences en réaffirmant la pertinence de l'avènement du couple régions-intercommunalités dans l'organisation des mobilités. Ainsi, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne pourront plus être AOM au-delà du 31 décembre 2020. les communes qui exerçaient précédemment leur compétence d'AOM et avaient constitué un réseau de transports publics en prélevant du versement transport devront transférer automatiquement cette compétence à leur EPCI. Toutefois, à titre d'exception, et pour des raisons géographiques, les communes dites isolées, c'est-à-dire les « îles » non membres d'un EPCI à fiscalité propre, pourront rester AOM sur leur territoire respectif. Par ailleurs, la disposition du projet de loi qui précise la possibilité pour les communes de transférer leur compétence à la communauté de communes à laquelle elles appartiennent- c'est l'alinéa 89 -devient superflue. Les communes sont déjà en mesure de transférer leur compétence. Quel

d'une rationalisation pour une meilleure visibilité, je ne partage pas tout à fait votre conclusion. À mon sens, ce que nos concitoyens attendent, c'est de l'efficacité et du service. Cela va d'un service de transport régulier ou du transport scolaire

ou d'accomplir un certain nombre de formalités. Le projet de loi vise à améliorer le service sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'il faut permettre, en accord avec les associations d'élus,

Vullien. L'article 1permet aux communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire aux communes « isolées » non membres d'un EPCI à fiscalité propre, de rester autorités organisatrices de la mobilité sur leur territoire.

Or, dans le cas où l'une de ces AOM choisit de ne pas exercer la compétence d'organisation du transport scolaire, le texte ne cible aucune collectivité chargée de cette mission. Afin de ne pas risquer une rupture de desserte scolaire sur ce territoire, cet amendement vise à faire en sorte que la région soit compétente pour organiser les services de transport scolaire à l'intérieur du ressort territorial de l'EPCI concerné.

avoir un consensus entre les différentes associations d'élus, qu'il s'agisse des communes, des intercommunalités, des régions ou des départements. Le

La création d'un nouveau cas de réversibilité nous fait revenir sur ce consensus. En tout cas, je peux vous l'assurer, les régions ne souhaitent pas qu'on introduise ce troisième cas de réversibilité ; cela crée une forme d'instabilité.

préciser le délai de trois ans. Il est prévu que les transferts interviennent à la demande de l'autorité organisatrice dans un délai convenu avec la région.

des lois. Nous avons souhaité introduire un cas supplémentaire de réversibilité fondé sur un commun accord entre la région et une communauté de communes. Il n'y a donc pas de transfert sans accord des deux parties. Notre

entre la région et une communauté de communes, on offrirait la possibilité à l'intercommunalité de reprendre la compétence. Il me semble très important, dans un esprit de dialogue- vous y avez fait référence -et d'intelligence territoriale,

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, qui a clarifié la répartition des compétences dans le domaine de la mobilité. Dans cette optique, notre amendement tend à prévoir que la prise de compétence en matière d'organisation de la mobilité par les communautés de communes s'effectue en un seul bloc, à l'exception des nouvelles compétences dévolues aux régions en application de la loi NOTRe : services non urbains, réguliers ou à la demande, et organisation des transports scolaires. Cet amendement vise à ne pas fragmenter la compétence mobilité afin d'éviter d'avoir deux autorités organisatrices responsables, pour des services différents, sur le territoire d'une même commune. Ainsi, en cas d'exercice de la compétence par la région, cette cohérence dans l'organisation des services sera également garantie. M. Patrick Chaize. L'alinéa 11 de l'article 1 du projet de loi d'orientation des mobilités n'autorise les communes à maintenir certains services qu'elles organisent déjà que dans les seuls cas où elles prélèvent le versement transport. Cette disposition manque de souplesse et ne correspond ni aux pratiques ni aux réalités du terrain. En effet, les communes qui assurent aujourd'hui des services de proximité à la demande ou d'accompagnement individualisé, par exemple, devraient pouvoir continuer à les offrir dans le cas où la région exerce la compétence en lieu et place de la communauté de communes dont elles sont membres, qu'elles aient ou non prélevé le versement transport avant le transfert.

n° 507 rectifié vise à clarifier une disposition du projet de loi prévoyant que les communes organisant déjà des services de mobilité pourront continuer à le faire lorsque la région deviendra AOM sur leur territoire. Cette faculté repose bien sur l'organisation de services et non sur leurs modalités de financement. L'amendement proposé permet d'éviter toute ambiguïté sur le dispositif. La commission a donc émis un avis favorable. Quant à l'amendement 340 rectifié, le projet de loi prévoit bien que chaque région devra assurer le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. Il ne nous paraît pas judicieux dès lors d'imposer par la loi les modalités de suivi du secteur des transports. Laissons les collectivités territoriales, une fois encore, se saisir de cette responsabilité

Dans ce contexte, les services de mobilité doivent pouvoir s'entendre comme l'ensemble des moyens concourant à la mobilité des personnes, qu'ils soient publics ou privés, collectifs ou individuels. Cet amendement vise donc à tirer les conséquences de cette approche au travers d'une définition élargie. est l'avis de la commission ? La portée de cet amendement est très incertaine et pourrait être source d'insécurité juridique. Par ailleurs, il ne revient pas aux AOM d'organiser de manière générale

et d'inscrire noir sur blanc que « les associations de représentants d'usagers, les personnels et leurs organisations syndicales, ainsi que les opérateurs en charge d'un service de transport public » participeront à la définition de cette offre, d'une part, pour des raisons démocratiques et, d'autre part, part, pour pouvoir bénéficier de leur expérience, voire de leur expertise, et de la pluralité des points de vue qu'il faut prendre en compte pour l'organisation des mobilités. Je pense à

Je pense aussi, à titre tout à fait personnel, à un collectif d'usagers de la ligne Paris-Granville qui fait en ce moment des propositions extrêmement pertinentes pour que le

connectée à la desserte TGV. Je pense enfin aux personnels et à leurs organisations syndicales qui possèdent eux aussi une expertise large et indiscutable dans l'organisation des transports : il s'agit non seulement de leur outil de travail, mais aussi de leur environnement.

Mme Christine Prunaud. La prise de conscience écologique générale pousse à imaginer de nouvelles solutions pour éviter le « tout-voiture » et à reconsidérer l'usage des transports collectifs. La transition écologique attendue de tous devra être inclusive et ne pourra pas se faire sur le dos des plus précaires. Inviter les automobilistes à abandonner leur voiture au profit des transports collectifs entreprise difficile, qui doit s'accompagner d'une politique tarifaire incitative. Beaucoup de villes ont déjà franchi le pas et il est temps de réfléchir de manière globale aux conséquences que pourrait avoir la gratuité totale ou partielle des transports en commun comme corollaire d'un droit au transport et à la mobilité.

Le Sénat se penchera sur le sujet dans le cadre d'une mission commune d'information demandée par notre groupe. Il faut Il faut d'ores et déjà ouvrir la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité d'en faire de même, d'autant que la gratuité s'envisage d'abord territoire par territoire, en fonction de l'état du réseau, du volume de passagers

de libre administration d'imposer à toute AOM d'engager des études sur un sujet spécifique, d'autant plus que, comme vous le savez, la gratuité des transports publics est un sujet qui fait largement débat au niveau national entre les différents acteurs du secteur. À ce jour, rares sont les AOM qui ont fait ce choix. La mission d'information créée récemment dans le cadre de l'exercice de son « droit

parce que je pense qu'il empiète sur les compétences des autorités organisatrices auxquelles il revient de fixer les tarifs. Ensuite, parce que la loi prévoit d'ores et déjà l'obligation de mettre en place des tarifs sociaux : la problématique mentionnée de l'accès au transport des publics fragiles est donc bien prise en compte et le projet de loi renforce la compétence des autorités organisatrices sur la mobilité solidaire. Au-delà de la question tarifaire,

liée au prix. Enfin, parce que, de façon générale, à un moment où beaucoup de nos concitoyens n'ont aucune alternative à la voiture individuelle, la priorité est de développer

transport est largement posée et suscite des positions très différentes alors même que chacun comprend

est à M. Guillaume Gontard. Dans un souci de préservation de l'environnement et de la santé publique, cet amendement vise à ajouter un objectif à l'action des autorités organisatrices de la mobilité. Elles devront ainsi favoriser le changement de pratique et le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives. Il s'agit simplement de préciser et d'expliciter ce que nous entendons par contribuer « aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l'air ». Il est inutile, mes chers collègues, que je vous refasse l'article sur l'usage des voitures individuelles. Rappelons tout de même que, sur l'ensemble des moyens de transport, les voitures particulières sont responsables de 54

Les nombreuses mobilisations de ces dernières années concernant les transports nous l'ont prouvé, nos concitoyens revendiquent plus de transports collectifs : plus de trains, des horaires étendus, l'extension et la modernisation des réseaux existants, la création de nouvelles lignes. De la même manière que l'attractivité des mobilités actives suscite un intérêt exponentiel, leur usage s'est largement démocratisé dans nos grandes villes. Il reste cependant insuffisant : 2 % seulement des Français se rendent au travail à vélo contre 31 % aux Pays-Bas ou, plus proche de nous, 5 % en Italie.

en raison non pas de freins individuels, mais d'un manque d'investissement public que nos concitoyens sont contraints à l'utilisation de leur véhicule personnel. Tout cela demande un investissement durable de la part de l'AOM en termes d'organisation, de coordination et de réflexion sur le partage des espaces. Les objectifs de lutte contre le changement climatique et la pollution de l'air doivent être clairement définis. C'est le sens de cet amendement que je vous invite tous, mes chers

La compétence d'organisation de la mobilité nouvellement dévolue aux régions s'accompagne d'une précision relative au périmètre sur lequel la région peut exercer ses missions. En effet, les services de mobilité pour lesquels la région devient compétente sont ceux « d'intérêt régional ». Or ce terme n'est pas précisément défini, ce qui risque d'engendrer des difficultés d'interprétation juridique. Le présent amendement tend donc à définir ces services comme ceux dont la mise en oeuvre opérationnelle n'est pas intégralement réalisée à l'intérieur du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ou d'un syndicat mixte de type « loi SRU » organisant, en lieu et place de ses membres, des services de transport publics réguliers ou à la demande. Quel

notamment dans une logique de rabattement vers une gare ou pour intensifier la desserte sur un territoire bien ciblé. J'ajoute que la notion d'intérêt régional est déjà utilisée dans le code des transports pour le transport ferroviaire et guidé, sans être définie. En souhaitant préciser certains points dans la loi, nous allons « verrouiller » le droit applicable et rendre impossibles des initiatives pourtant tout à fait pertinentes et utiles au niveau local. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

en matière d'organisation des mobilités à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à une autre autorité organisatrice de la mobilité.

constateraient un besoin de mobilités non satisfait dépassant leurs propres ressorts territoriaux. Nous considérons que cette possibilité donnée aux AOM est importante en ce qu'elle permet de signaler les

de supprimer les zones blanches de la mobilité dénoncées par Mme la ministre. C'est la raison pour laquelle nous proposons de réintroduire cette possibilité en cas de délégation permettant de répondre aux besoins de mobilités des territoires.

présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.

n'emportent ni diminution des ressources publiques ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions posées étant à la seule charge des opérateurs. Voilà qui est fait pour rassurer.

En présence de droits spéciaux ou exclusifs d'exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d'autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s'agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme au plus tard le 31 décembre 2024, comme le prévoit le code des transports, dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d'exclusivité qu'ils contiennent. Un avis conforme préalable du gestionnaire de voirie a pour objet de prendre en compte ces contraintes, notamment en ce qui concerne le lieu et l'implantation des points d'arrêt, mais aussi au regard de considérations y afférentes, notamment liées à la maîtrise des risques de congestion des voies. Cet amendement, en ce qu'il a pour objet de préciser les conditions d'exploitation des services de transports à vocation touristique, n'emporte ni diminution des ressources publiques ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.

qu'ils contiennent. Un avis conforme préalable du gestionnaire de voirie a pour objet de prendre en compte ces contraintes, notamment en ce qui concerne le lieu et l'implantation des points d'arrêt, mais aussi au regard de considérations y afférentes, notamment liées à la maîtrise des risques de congestion des voies. Cet amendement, en ce qu'il a pour objet de préciser

C'est le monde rural qui défend un amendement parisien ... À Paris, l'exploitation des lignes régulières à vocation touristique relève d'une double compétence : celle de l'autorité organisatrice des services Mobilités, mais aussi celle de la Ville de Paris en tant que gestionnaire de domaine pour la définition des conditions de circulation et la gestion des points d'arrêt. Il est proposé de définir ce double niveau de compétence pour permettre une croissance maitrisée de ces lignes.

d'organiser les transports à vocation touristique lorsqu'ils constituent des services publics réguliers. Ces six amendements vont dans le même sens, en apportant différentes précisions à ces dispositions.

à permettre à toutes les autorités d'intégrer des prescriptions environnementales dans leur cahier des charges, après avoir obtenu un avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie, et à préserver des conventions existantes à la date d'entrée en vigueur du présent

En effet, en matière de gabarits routiers, l'État applique des critères indifférenciés sur les infrastructures où il est maître d'ouvrage, avec des portions en 2x2 voies souvent trop chères et inutiles du fait de la faible fréquentation dans les territoires ruraux. L'idée est donc de permettre de passer à des gabarits moins imposants, mais plus faciles à financer, ce qui contribuerait à la mobilité et au désenclavement des territoires.

qui ont vocation à aborder la planification régionale des infrastructures de transport. Par ailleurs, aucune norme n'impose à l'État de surdimensionner ses projets sur des territoires qui ne le nécessiteraient pas.

la métropole du Grand Paris, née en 2016, n'y dispose encore d'aucun siège. Le présent amendement a pour objet d'actualiser la composition du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités en y intégrant un siège pour la métropole du Grand Paris, Paris Île-de-France et les autres EPCI d'Île-de-France, c'est-à-dire sans modifier la composition de l'établissement public. Un décret en Conseil d'État sera nécessaire pour en tirer les conséquences sur le nombre total de sièges et leur répartition. L'amendement

Olivier Léonhardt. En Île-de-France comme dans de nombreuses régions de notre pays, la répartition des investissements en matière de transports entre les coeurs d'agglomération et les zones périurbaines est souvent très déséquilibrée. Les Franciliens qui vivent dans les départements de la grande couronne et qui utilisent les transports en commun subissent chaque jour les conséquences de trente

contre un peu moins de la moitié de ce temps pour les habitants de la zone très dense. Ils subissent, par ailleurs, des conditions de transport bien plus inconfortables. Le réseau existant est au bord de l'implosion : trains supprimés ou bondés, affaissement des voies, retards, lignes fermées sont leur quotidien. Ce déséquilibre dans les investissements est d'autant plus dommageable que ce sont les habitants des zones périurbaines qui utilisent, parce qu'ils y sont contraints, leur voiture. C'est à eux qu'il faudrait offrir une alternative si nous voulons réduire la pollution.

Cette situation ubuesque est due, pour partie, à la gouvernance totalement déséquilibrée d'Île-de-France Mobilités. J'ai donc déposé plusieurs amendements pour rectifier cette situation. La Ville de Paris est surreprésentée par rapport aux autres départements, ce qui n'est justifié ni par son financement ni par son nombre d'habitants. Elle dispose de cinq sièges, quand les autres départements n'en ont qu'un seul. Les principaux financeurs- les entreprises, avec le versement transport -ne disposent que d'un siège sur vingt-neuf, et les usagers, deuxième financeur d'Île-de-France Mobilités,

Toutes les régions sont concernées par ces déséquilibres. Je voudrais donc faire appel à la solidarité des collègues des territoires périurbains de toutes les régions : associons les usagers

par ailleurs présidente d'Île-de-France Mobilités, s'était déclarée opposée à l'intégration d'un siège pour la métropole dans le conseil administration. En effet, ce sont en réalité les départements franciliens qui ont des compétences en matière de voirie et qui sont à ce titre représentés.

prenantes, mais un lieu de décision. Les usagers sont pleinement représentés au sein du comité des partenaires d'Île-de-France Mobilités, qui sert d'ailleurs d'exemple dans le présent projet de loi pour généraliser cette instance auprès de chaque autorité organisatrice.

La logique du système actuel est que la région, la Ville de Paris et les départements franciliens sont membres d'Île-de-France Mobilités parce qu'ils lui apportent également des financements, de l'ordre de 1,3 milliard d'euros par an. par an. Cette réflexion sur la place de la métropole du Grand Paris au sein du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités ne peut pas être menée indépendamment d'une réflexion plus globale sur la gouvernance et le financement des transports en Île-de-France. L'amendement n° 691 rectifié me semble prématuré par rapport à cette réflexion.

et le poids des différents départements, et le poids de la Ville de Paris sont liés aux clés de financement. La part des collectivités représente 20 % du financement d'Île-de-France Mobilités, près de 50 % étant assurés par les entreprises au travers du versement transport. Parmi les collectivités, la représentation est faite au prorata des contributions de chacun. De façon générale, la consultation des usagers

est de permettre à l'autorité organisatrice des services de transports scolaires d'ouvrir ses services à d'autres usagers : travailleurs, personnes isolées, retraités.

mais la mesure proposée permet d'envoyer un signal favorable à cette pratique qui améliore effectivement la desserte des territoires ruraux par des services de transport public, là où l'organisation de nouveaux services réguliers aurait un coût excessif. L'avis est donc favorable,

pour apporter, par exemple, un surcroît de desserte en faveur de leurs habitants. Quant au principe d'une ouverture des services de transport scolaire à des personnes tierces, l'amendement n° 510 que nous nous apprêtons à adopter permet de réaffirmer cette perspective. je demande le retrait l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires à ouvrir ces services à d'autres usagers. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, cet amendement est déjà satisfait puisque les autorités organisatrices peuvent déjà choisir d'accueillir dans les services de transports scolaires d'autres publics dans l'optique d'une politique de mutualisation. Elles doivent le faire en prenant en considération l'opportunité de mutualiser et la capacité des cars aux horaires de ramassage scolaire. Elles doivent aussi veiller au maintien de la vocation scolaire du service, ainsi qu'aux obligations afférentes en matière de sécurité. Je suis convaincue qu'il s'agit d'une très bonne base pour structurer des services dans des territoires où, bien souvent, les transports scolaires sont le seul transport régulier ; mais le droit le permet déjà. J'émets donc un avis de sagesse sur l'amendement n° 510. Pour les mêmes raisons,

communautés de communes ou régions, qui auront pour mission de coordonner les modes de déplacement sur leur territoire. C'est pourquoi je vous propose d'instaurer une consultation obligatoire des autorités organisatrices par les établissements scolaires lors de la modification des horaires ou de la carte scolaire, afin de favoriser le décalage des horaires d'entrée et de sortie de ces établissements pour permettre d'enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur. Cette mesure présente plusieurs avantages pour les collectivités en charge du transport scolaire. Elle permettrait de faire des économies en réalisant autant de circuits avec moins de véhicules de véhicules ; de baisser le nombre de véhicules en circulation, ce qui diminue d'autant les émissions polluantes ; enfin, d'améliorer les conditions de travail des conducteurs, souvent employés à temps partiel, qui verraient leur temps de travail allongé. Cette proposition se veut

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré la compétence des transports interurbains et scolaires aux régions. Depuis 2016, celles-ci ont donc de nouvelles attributions, qui nécessitent notamment une coordination avec le ministère de l'éducation nationale. Cet amendement tend à ajouter dans le code de l'éducation une procédure de consultation des autorités organisatrices par les représentants de l'éducation nationale, afin de favoriser le décalage des horaires d'entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre d'enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur. Cette mesure présente plusieurs avantages pour l'ensemble des acteurs. Les collectivités territoriales pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service. Cette mesure produirait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation. Elle permettrait enfin l'emploi des conducteurs sur des durées de travail plus longues, par exemple avec deux circuits au lieu d'un.

probablement plus complète pour ce qui concerne la mise en place de modalités de consultations entre les régions organisatrices et le ministère de l'éducation nationale. C'est la seule petite différence que je tenais à souligner.

? Je précise que des dispositions réglementaires existent déjà dans le code de l'éducation sur les modalités de consultation des AOM quant aux changements d'organisation,

Une meilleure articulation des horaires scolaires peut permettre d'optimiser des services de transports scolaires

pour les conducteurs de ces cars. Je confirme que ces dispositions sont d'ores et déjà codifiées à l'article D. 213-29 du code de l'éducation. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, cet article n'a pas été

du quotidien. Les transports du quotidien peuvent être définis comme les services de transport de voyageurs d'intérêt économique général offerts au public, sans discrimination et en permanence, ce qui correspond, en France, au service de transport conventionné, c'est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Il est donc primordial que les transports publics du quotidien soient désormais considérés comme un service de première nécessité- personne ne peut, me semble-t-il, en disconvenir -, comme ils le sont d'ailleurs déjà chez nos voisins européens que sont la Belgique, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, le Portugal ou le Royaume-Uni, et qu'ils bénéficient de fait d'un taux de TVA

de l'accès aux transports et aux mobilités d'une certaine partie de la population. Nous savons combien est fondamental le rôle du transport public de voyageurs pour favoriser la mobilité de tous et lutter contre toute forme d'exclusion, notamment pour faciliter l'accès à l'emploi.

que nous avons eus en 2013 lors de l'augmentation des différents taux de TVA, pour financer le fameux CICE ... Je me souviens notamment de la réponse du ministre Hamon lorsque je l'avais interrogé sur ce sujet : il disait que le CICE allait grandement profiter aux entreprises du secteur du transport cela compenserait la hausse de TVA. Six ans plus tard, les faits démontrent qu'il n'en a rien été et nous donnent fortement raison. Depuis 2014, le taux intermédiaire qui s'applique aux transports est donc passé de 7 % à 10 %.

tous et toutes demandent un taux réduit à 5 % pour les transports publics. Cette proposition de baisse de la TVA est une mesure de bon sens, puisque les transports publics participent aux objectifs de transition énergétique et ont un rôle social de première utilité. Je me permets d'ailleurs de rappeler que les transports publics sont classés classés comme tels en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal, en Suède ou encore en Norvège. On cite souvent ici les exemples européens ; à notre tour de rappeler à notre Haute Assemblée comment les choses se passent chez nos voisins. Aussi, à l'heure où la jeunesse se mobilise au plan mondial en faveur du climat et où le Gouvernement entend avec ce projet de loi « révolutionner » les mobilités, voter cet amendement irait dans le bon sens. Même à cette heure tardive, j'espère avoir gagné l'appui de mes collègues,

Je souscris au fait que les transports, plus que jamais aujourd'hui, à l'heure où les inégalités sont si fortes dans ce domaine, comme cela s'est exprimé depuis quelques mois, sont un service de première nécessité. Néanmoins, la rédaction pose des difficultés de périmètre- comment définit-on les transports publics de voyageurs du quotidien ? -, de coût

nous avons déjà eu ce débat à l'occasion du pacte ferroviaire. Aux termes de votre amendement, ma chère collègue, le taux réduit de TVA s'appliquerait aux transports publics soumis à des obligations de service public, comme les TER et les TET. Mais, en réalité, la demande de ce taux réduit concerne également les transports urbains, ceux qui desservent aussi des zones rurales où il est aujourd'hui difficile d'organiser du transport public régulier. L'application d'un tel taux réduit devrait être plus globale, car les transports sont, comme je viens de le dire, aujourd'hui plus que jamais, un service de de première nécessité. Mais il n'est pas facile aujourd'hui de délimiter clairement le périmètre qui pourrait être concerné, et les montants mis en jeu seraient évidemment très importants. Nous avons tenté en commission

Le scrutin est ouvert.

Cet amendement vise à doter les collectivités territoriales d'un nouvel outil facultatif pour contribuer à financer de grandes infrastructures. Des dispositifs proches existent dans de nombreux pays, pas dans le nôtre. Autour d'une gare TGV ou d'un arrêt de tramway, par exemple, on constate très régulièrement des augmentations très nettes des valeurs immobilières.

pour les logements anciens, nous proposons de majorer les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière d'un maximum de 0,5 % pour une durée limitée et prédéterminée.

Ces difficultés demeurent, alors même que 85 % des Français résident à moins de cinq kilomètres d'un service public ou d'un mode de transport. En outre, ces politiques de transports induisent des modes de déplacement énergivores et participent à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en 2017, les transports en France étaient responsables de près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre et de 38 % des émissions de CO2. De même, plus de la moitié des émissions de CO2 des transports provient des voitures particulières. Or la situation climatique et les objectifs fixés par l'accord de Paris nous commandent de modifier nos habitudes et de repenser en profondeur notre rapport à la mobilité et aux modes de déplacement. Le développement des mobilités actives aura également des effets positifs en matière de santé publique. Selon une étude du Commissariat général au développement durable de mai 2016, le développement de l'usage du vélo et des transports en commun présenterait un bilan positif de plus d'un milliard d'euros. Ainsi, le présent amendement vise à reconnaître à chaque personne la possibilité d'utiliser un mode de transport actif afin de relier, dans des conditions sécurisées, son domicile et son lieu de travail, ainsi que les lieux offrant des services publics et non publics situés à de courtes distances. Pour les plus grandes distances, la multimodalité doit permettre, dans un grand nombre de situations, d'intégrer la mobilité active pour une partie du trajet à parcourir. Je rappelle que 75 % des déplacements quotidiens font moins de huit kilomètres et que la notion de courte distance concerne tous les déplacements inférieurs à dix Afin de rendre cet objectif effectif, l'État et les collectivités locales en charge des politiques de transport doivent prendre des mesures adéquates, notamment à travers l'éducation des plus jeunes, la sensibilisation des adultes à l'usage du vélo, à l'utilité des trajets à pied sur de petites distances, ainsi qu'à la sécurisation de ces modes de transport, afin d'encourager leur usage.

d'itinéraires cyclables, par la lutte contre le vol des vélos- avec le marquage des vélos et le développement de garages sécurités-, par la mise en place d'un forfait mobilité durable et par l'apprentissage du vélo- à travers le

bis Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 116 amendements au cours de la journée, dont 78 ce soir ; il en reste 661 à examiner sur ce texte.